Monsieur le président,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

dû interrompre nos travaux à l'article 21 sans pouvoir poursuivre nos débats. Il nous reste donc 440 amendements à examiner d'ici à demain soir, ce qui représente un volume

nous avons 303 amendements à examiner sur la fiscalité écologique et environnementale. Enfin, le Gouvernement ayant déposé plusieurs amendements la nuit dernière,

Selon l'article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

La séance est suspendue.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article traditionnel vise à fixer le montant de la Je tiens à le souligner, comme l'aurait fait à ma place M. Raynal, la stabilité globale des dotations pour nos collectivités est un premier pas. Cependant, cette situation n'est pas optimale pour elles, et ce pour deux raisons sur lesquelles je souhaite interpeller le Gouvernement. En premier lieu, c'est la question de la réforme de la DGF, initiée durant le quinquennat précédent avec les travaux de notre regretté collègue Jean Germain et de Christine Pires Beaune, députée. Quand le Gouvernement va-t-il enfin se décider à poursuivre ces travaux pour achever ces réformes, en particulier la révision des valeurs locatives, qui concerne énormément de logements

lieu, dans l'attente de cette réforme, il faudra que nous nous mettions d'accord sur ce que l'on entend par « stabilité des dotations », car les collectivités- et on ne peut pas vraiment les en blâmer -ne semblent pas avoir la même lecture que celle qui est proposée par le Gouvernement. C'est tout d'abord la non-indexation sur l'inflation qui fait sujet. Il en est de même de la progression de la péréquation plus précisément, vous le savez, nous sommes favorables à la montée en puissance des mécanismes péréquateurs, mais non pas par le biais de l'écrêtement, comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin, se pose la question des variables d'ajustement : sur le plan symbolique, reprendre de la main droite ce que l'on donne de la main gauche ne me paraît ni lisible ni efficace. En clair, si cet article est moins sévère qu'on a pu constater dans les exercices antérieurs- il faut bien l'avouer -, je ne pense pas qu'il faille pour autant donner un blanc-seing au Gouvernement, car, au quotidien, ce sont nos services publics locaux qui subissent cette logique étatique de réduction continue du financement de la vie de nos territoires. La parole

on devait faire avec 139 euros par habitant de DGF ; l'année dernière, on était à 13 euros par habitant de DGF ; demain, on sera à 0 euro par habitant de DGF. Et je ne parle même pas de certaines communes de mon département qui, aujourd'hui, ne perçoivent plus de DGF, se voient même appliquer une contribution au redressement des finances publiques, et donc donnent de l'argent à l'État sur leurs recettes. Elles sont à taux négatif ! C'est fantastique : si l'État faisait pareil, on n'en serait pas à ce niveau d'endettement ! Comme je connais le sort qui va être réservé à ces amendements et puisque nous sommes pressés, je les retire.

Cela ne semble pas équitable au regard des défis auxquels font face les territoires ruraux en termes d'attractivité, d'activité économique et de démographie. Aussi, afin de permettre à la ruralité et à l'hyper-ruralité de rattraper leur retard, il convient de doter la DSR d'un montant équivalent à celui de la DSU. Les mécanismes actuels de péréquation et les moyens financiers qui sont alloués sont insuffisants. Dans ce but, le présent amendement vise à revaloriser le montant de la DGF d'environ 600 millions d'euros, lequel sera réparti entre les différentes dotations de péréquation

pour pouvoir recevoir leur courrier- cela répond à un besoin minimum de dignité -et effectuer un très grand nombre de démarches. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sans domicile peinent à accéder à ce service ; en effet, de nombreux CCAS ou CIAS sont saturés

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, l'Assemblée nationale a modifié les critères de potentiel financier permettant l'éligibilité à cette dotation Natura 2000, de sorte que, en 2020, davantage de communes seront éligibles.

Pour rappel, l'article 15 de la loi de finances pour 2016 a institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant aux AOM la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Ce prélèvement s'élevait à 90,6 millions d'euros en loi de finances pour Le Gouvernement se félicite de cette « innovation », en soulignant qu'elle « permet d'alléger l'effort de maîtrise de la trajectoire des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, reposant sur les variables d'ajustement ». Concrètement, le Gouvernement diminue quasiment de 50 % la dotation de compensation VT pour pour faire participer les collectivités territoriales elles-mêmes au financement, au profit des régions, de la réforme de l'apprentissage- 72 millions d'euros -, de la progression des dotations de soutien à l'investissement local- pour un montant non précisé dans les documents budgétaires -, de la progression du montant des compensations fiscales- 123 millions d'euros -, de la hausse du prélèvement sur recettes de l'État versé la hausse de la dotation élu local, liée au projet de loi Engagement et proximité- 10 millions d'euros -, de la hausse de la dotation pour les titres sécurisés- 6 millions d'euros -, de l'abondement du fonds d'aide au relogement d'urgence- 1,5 million d'euros. Le principe de l'enveloppe normée pour les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales finit par être mortifère. Face à des variables d'ajustement au plus bas, le Gouvernement cherche des des lignes à minorer au sein de cette enveloppe. Nul doute que les mécanismes de compensation résultant de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales entreront à terme dans ce champ. L'amendement

Cette minoration devait servir à financer plusieurs mesures, notamment la suppression des indemnités de conseil aux comptables publics versées par les collectivités territoriales, soit 25 millions d'euros. Or, en réalité, cette prise en charge financière, initialement imposée aux communes, servirait surtout à financer la réforme du réseau des trésoreries ; ce qui demeure scandaleux. La suppression des indemnités de conseil s'inscrit bien évidemment dans le bon sens. En effet, l'administration fiscale ne peut être rétribuée pour des missions de conseil faisant partie de ses missions. À l'heure des réductions drastiques de la dotation globale de fonctionnement et des difficultés financières rencontrées par les communes, le versement d'une indemnité de conseil au receveur du Trésor public ne paraît ni nécessaire ni légitime. Surtout, il convient de préciser que la demande d'indemnisation pour de tels conseils, à laquelle la collectivité demeure libre de souscrire ou non, peut s'appliquer sur tous les budgets : communaux, intercommunaux, annexes, etc. Cela demeure profondément choquant. De plus, ces « étrennes » laissent planer sur la collectivité une sorte de pression quant à l'implication, dans le futur, du receveur. Plusieurs collectivités ont d'ailleurs déjà voté des baisses ou la fin de cette mesure. Alors que la prévention des conflits d'intérêts est au coeur des politiques publiques, ce procédé ne peut plus durer. Néanmoins, il n'est pas acceptable que l'État fasse supporter par les communes ce que lui-même doit prendre en charge. Ces modifications n'ont en aucun cas à être financées par les collectivités territoriales : ces dernières n'ont pas vocation à être les victimes collatérales. C'est pourquoi le présent amendement prévoit, notamment, de remettre à la charge de l'État le coût de cette mesure.

la question de la confiance entre l'État et les collectivités locales. Le Gouvernement et le Président de la République font des efforts pour essayer de retisser le lien avec les collectivités. Dans ce contexte, j'aimerais que vous changiez de discours sur un point : je veux que vous réaffirmiez que vous continuez à demander aux collectivités locales de faire des efforts.

effet, il s'agit de voter les transferts financiers aux collectivités territoriales, soit plus de 115 milliards d'euros,

Alors, quand j'entends qu'il faudra aussi mettre à contribution les départements et les régions pour payer les indemnités des maires, franchement, ce n'est pas admissible

Delcros. Le présent amendement concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2011, ces fonds sont alimentés par une dotation faisant l'objet d'un prélèvement sur les recettes de l'État.

Mon amendement vise à rétablir, sous forme de prélèvement sur recettes (PSR), la somme de 27 millions d'euros attribuée cette année à la collectivité territoriale de Guyane

La collectivité a effectivement bénéficié, jusqu'en 2016, de la dotation globale garantie correspondant aux ressources de l'octroi de mer. À compter de l'exercice 2017, et de façon progressive, le produit de l'octroi de mer a été transféré aux communes guyanaises, comme dans les autres territoires ultramarins. Cette perte de ressources pour la collectivité territoriale de Guyane a fait l'objet d'une compensation pour les exercices 2017, 2018 et 2019, à proportion des transferts effectués aux communes, sous la forme d'un PSR. Ce dernier s'élève, en 2019, à 27 millions d'euros. Le présent projet de loi de finances, au sein de son article 21, transforme ce prélèvement sur recettes en une dotation dans le montant ne peut excéder 27 millions d'euros. Cette évolution est particulièrement préoccupante puisque le PSR correspondait à un engagement du Gouvernement à maintenir une compensation égale à 27 millions d'euros en 2019, et au-delà.

Produit des compensations d'exonérations de taxe sur le foncier bâti accordées par l'État en 2019 : 11 865 euros ! Donc, pour 600 logements exonérés de taxe sur le foncier bâti, l'État verse 11 865

Lavarde. Je reviens sur un sujet déjà abordé lors de l'examen du PLF pour 2017, à savoir les coûts liés aux transferts successifs de charges d'état civil prévus notamment par la loi de modernisation de la justice du XXI siècle.

perçue par la Polynésie française, le projet de loi de finances pour 2020 transforme en prélèvement sur recettes la DGA jusqu'ici inscrite à titre indicatif sur le programme 123, Conditions de vie outre-mer, de la mission " Outre-mer " du budget général.

républicain avaient alors alerté sur la dangerosité et l'inconstitutionnalité de ce changement de règle. Le Gouvernement n'avait rien voulu entendre, mais le Conseil constitutionnel nous a donné raison en censurant la mesure.

après cette date. Pourtant, le montant pris en compte au titre de la compensation financière par le département des dépenses transférées à l'État comprend déjà des rappels. L'alinéa 109 fait donc supporter au département deux fois le coût de ces rappels : il est indispensable de le modifier.

Ce fonds vise à accompagner le financement par les départements des allocations individuelles de solidarité- RSA, APA, et PCH -par voie de péréquation horizontale, et donc sans accroissement de la charge budgétaire de l'État.

et de Martinique dans le cadre de croisières maritimes. Ce dispositif vise à renforcer la compétitivité de ces territoires et à y développer le commerce local. Il est demandé de longue date par les acteurs locaux, et pour cause : dans les autres États de la Caraïbe, l'exemption totale de taxes est presque toujours la règle. Ce dispositif met en oeuvre la mesure 39 présentée dans le cadre du conseil interministériel de la mer du 17 novembre 2017.

en oeuvre, à titre expérimental, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes de croisière accostant en Martinique ou en Guadeloupe. Plusieurs dizaines de milliers de croisiéristes font étape chaque année dans ces collectivités, mais ils dépensent très peu dans les centres-villes qu'ils visitent, en raison du coût relativement élevé

au moins les compagnies maritimes et les compagnies aériennes, qui sont exonérées d'octroi de mer et de TICPE pour le gazole et le fioul lourd,

Michel Magras. Cet amendement vise à élargir le champ du crédit d'impôt ouvert aux organismes d'habitation à loyer modéré en outre-mer, afin d'encourager la réalisation des travaux de désamiantage, de réhabilitation ou de démolition des logements achevés depuis plus de vingt ans. Le parc locatif existant, déjà insuffisant au regard des besoins, se caractérise en outre par sa vétusté. Tout en fixant dans la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer un objectif ambitieux

de nombreux logements révèlent la présence d'amiante, comme en atteste la réalisation d'une étude sur le développement de filières amiante outre-mer. Le présent amendement vise donc également à introduire une incitation à la démolition, afin qu'elle soit privilégiée lorsqu'elle s'avère plus économique

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Merci